que les décisions de la commission départementale, qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant leur publication, ne peuvent pas être ultérieurement contestées à l'occasion d'un recours contre les impositions établies à partir des tarifs fixés par la Commission

Le présent amendement vise à garantir que les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties arrêtés par la commission départementale ne puissent être contestés que par la voie de l'action dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Cette solution est conforme à ce que la loi et la jurisprudence prévoient respectivement, s'agissant des recours contentieux ouverts à l'encontre des tarifs d'évaluation applicables aux propriétés bâties et aux locaux professionnels. Dans ces conditions, la commission spéciale est favorable à cet amendement. La parole

compatibles avec l'organisation souhaitée par le Gouvernement, qui propose de confier les missions de l'observatoire à la cellule du bâti scolaire rattachée au secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Nous ne minimisons pas

dans cette cellule. Quel est l'avis de la commission spéciale ? La volonté du Gouvernement de supprimer l'Observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement a de quoi surprendre. En février 2019, c'est pourtant lui qui introduisait, par un amendement au projet de loi pour une école de la confiance, une disposition obligeant les collectivités territoriales à suivre les recommandations de cet observatoire pour la construction ou la rénovation de tout bâtiment scolaire. C'est bien le signe qu'il jugeait alors les travaux de cet observatoire importants et précieux. Dès lors, comment expliquer un tel revirement ? À la différence d'autres organes mentionnés dans ce texte, cet observatoire fonctionne bien : il a tenu près de soixante-dix réunions en 2018. Le très grand nombre d'acteurs qu'il mobilise, présenté comme un handicap par le Gouvernement dans son argumentaire, n'est donc pas un problème. Au contraire, un tel fonctionnement permet de prendre en compte la diversité des parties prenantes. En outre, le bâti scolaire En outre, le bâti scolaire relève de la compétence des collectivités territoriales depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avaient justifié la création de cet observatoire en 1995. J'ai interrogé les services de l'État sur la manière dont ils comptaient associer les collectivités territoriales sur ces sujets à l'avenir.

d'État. Le présent amendement répond au souhait du Gouvernement de supprimer la Commission scientifique nationale des collections, qui avait été créée par l'article 4 de la loi du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections. Cette instance dédiée au déclassement, qui n'a eu à traiter que peu de demandes en la matière puisqu'elle a rendu huit avis en cinq ans, a achevé le travail doctrinal que lui avait confié le législateur. Ce travail s'est matérialisé par l'élaboration d'un rapport assorti de recommandations, remis au Parlement en 2015. Contrairement à certaines craintes ou interprétations, la suppression de cette commission n'emporte pas d'effet sur l'intégrité des collections publiques et leur inaliénabilité : cette commission rendait uniquement un avis sur les propositions de déclassement du domaine public, ce qui supposait de faire le constat de la perte d'intérêt public des biens des biens concernés. Elle n'avait nullement été dotée des compétences nécessaires pour traiter les cas de restitutions internationales, comme celles qui sont envisagées pour le patrimoine africain. Ces restitutions, qui nécessitent de procéder à une sortie des collections publiques, ne reposent pas sur le constat de la perte d'intérêt public des biens concernés, et se différencient donc du déclassement administratif. Elles impliquent par ailleurs nécessairement de passer par une mesure législative. La décision de déclassement du domaine public, qui relève d'une procédure administrative, continuera de se fonder sur la justification d'un rapport argumenté,

puisse se prononcer sur les décisions de déclassement des biens culturels appartenant aux collections publiques. Cette procédure constitue une garantie qu'aucune atteinte excessive n'est portée au principe d'inaliénabilité Il serait incohérent de la supprimer, alors même que toute entrée d'un bien dans les collections est, de son côté, soumise à l'avis préalable d'instances scientifiques. Le bilan de cette commission n'est pas négligeable, qu'il s'agisse de l'élaboration d'une doctrine en matière de déclassement ou de la réflexion sur la question sensible des restes humains. Son maintien est pleinement justifié, mais il faut la rendre plus agile et plus réactive. Rien n'empêcherait aujourd'hui le pouvoir réglementaire de remédier à ses difficultés de fonctionnement en réduisant le nombre de ses membres et en supprimant les différents collèges. La commission spéciale

à des juristes, des scientifiques, des philosophes, à toutes personnalités susceptibles d'éclairer le politique pour éviter certaines lois de circonstance n'ayant pas lieu d'être,

de ces objets et de la façon dont on peut ou non les restituer. L'administration de la culture a très finement joué en créant une commission qui ne pouvait pas

Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Je voudrais cependant apporter deux éléments au débat. Premièrement, la commission dont nous proposons la suppression n'est pas compétente en matière de restitutions.

le Parlement sera de toute manière appelé à se prononcer sur toute forme de restitution, puisque la restitution déroge au principe législatif d'inaliénabilité des collections. Par ailleurs, le déclassement

que sa suppression n'interdirait évidemment pas au Parlement d'être éclairé par les travaux des différents acteurs et des services de l'État, sachant que,, le Parlement, et donc le peuple français, aurait à se prononcer sur toute forme de restitution. L'ensemble de ces éléments m'amènent à maintenir cet amendement,

Cette commission nationale n'a pas les mêmes missions que les délégations aux outre-mer qui ont été créées par la suite à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Alors que nos compatriotes d'outre-mer sont trop souvent relégués au second plan par les politiques gouvernementales,

L'intention de leurs auteurs est pleinement compréhensible, et je partage naturellement leur souci de l'efficience des politiques de l'État dans ces territoires spécifiques que sont les outre-mer.

particulier. Son rapport biennal 2018-2019 n'aborde toutefois ces sujets qu'incidemment ; autrement dit, elle ne suit plus les priorités qui lui ont pourtant été données par le législateur. Je rappelle que ces missions restent à l'inverse pleinement exercées par les délégations parlementaires aux outre-mer.

François Bonhomme, pour explication de vote.

explication de vote. Je vais essayer, à cette heure tardive, de ramener un peu de sérénité dans notre hémicycle.

secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d'abroger la section du code de l'environnement relative à l'existence et au fonctionnement de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs

Elle ne s'est ensuite réunie qu'une dizaine de fois entre 2011 et 2012 ; à l'issue de cette période, elle a produit un rapport public, constatant qu'elle ne bénéficiait que d'une faible implication du Parlement et faisant état de ses réserves sur sa propre capacité à fonctionner de manière pérenne. En tout état de cause, la CNEF ne s'est plus réunie depuis 2012. Le rapport faisait également état du manque de moyens humains mis à sa disposition, en comparaison de l'affectation de moyens humains très importants- une quinzaine de rapporteurs et l'assistance d'un groupe d'experts -à la rédaction du rapport de la Cour des comptes de 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire, un rapport mis à jour en 2014. des comptes a par la suite continué à examiner en profondeur la question de la prise en compte des coûts de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, dans son rapport de juillet 2019 sur l'aval du cycle du combustible nucléaire,

À ce jour, la CNEF est en droit le seul organe mixte comprenant des parlementaires et informant le grand public dans le domaine du démantèlement des installations nucléaires Par ailleurs, le contexte de la transition énergétique est peu propice à la suppression de la CNEF. Tout d'abord, depuis la promulgation de la loi Énergie-climat de 2019, l'article L.

et du provisionnement des charges afférentes se pose donc avec plus d'acuité encore que lors de l'institution de la CNEF, en 2006. La Cour des comptes estime d'ailleurs que ce provisionnement pourrait renchérir le coût de l'énergie nucléaire. Dans son rapport de 2014, elle appelle non pas à supprimer la CNEF, mais à en repenser « le rôle, le positionnement et la composition ». C'est pourquoi la commission spéciale n'a pas souhaité supprimer la CNEF, préférant engager sa revitalisation en lui permettant de saisir l'ACPR.

à la hauteur des opérations de démantèlement à venir. Il paraît tout à fait essentiel qu'un tel suivi puisse être effectué en toute indépendance, sous le contrôle du Parlement. C'est le cas avec cette commission à la

présentant cette évaluation, qui est rendu public. Elle peut aussi adresser à tout moment des avis au Parlement et au Gouvernement. Ces rapports décrivent l'évaluation des charges, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges, les choix retenus concernant la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions. La CNEF peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Pour ces raisons, nous ne pensons pas qu'il soit opportun de supprimer cette commission,

Jean-Paul Émorine, pour explication de vote.

quant aux conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 232 de la loi de finances pour 2019, qui visent à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie trouve sa cause dans les essais nucléaires. Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de la double reconnaissance des victimes des essais nucléaires français et de leur droit à indemnisation. Il vise à ajuster le dispositif d'indemnisation des maladies dues aux essais nucléaires. Pour mémoire, en novembre 2018, une commission associant parlementaires et personnalités qualifiées, chargée de faire toutes propositions propres à consolider la procédure d'indemnisation, a fait le choix d'une indemnisation intégrale fondée sur le critère d'une dose maximale admise pour le public par la législation française et sur les bases des règles européennes et des recommandations internationales. Nous voulons, au travers de cet amendement, sécuriser la mise en oeuvre de ces dispositions

est de coordonner l'accompagnement médical des riverains français des essais ayant été effectués en Algérie et en Polynésie entre 1945 et 1995.

Depuis 2012, la représentation du secteur mutualiste est assurée au sein du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), dont la mission est de donner un avis sur tous les projets de textes normatifs traitant des questions relatives à l'assurance ou au secteur mutualiste. Depuis cette date, les projets de textes relatifs à la mutualité

Par ailleurs, le CSM est également chargé de présenter toute suggestion concernant la mutualité ou les bonnes pratiques applicables à ce secteur. En réalité et en pratique, il est très peu actif sur ce point, puisque la commission plénière ne s'est réunie que trois fois depuis 2012, essentiellement pour examiner des nominations de membres de commissions spécialisées.

Je précise que le CSM est chargé d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, par le biais d'une commission spécialisée. Ce fonds attribue des prêts et des subventions aux mutuelles qui ont une activité d'oeuvre sociale. Si cette mission du CSM est supprimée, il n'est pas pour autant question de supprimer ledit fonds.

Il ne vous aura toutefois pas échappé que le sujet des mutuelles est extrêmement sensible dans la vie sociale de ce pays. Vous avez fait état d'un certain nombre de questions de procédure, mais la réalité, vous le savez, est que le mouvement mutualiste dans son ensemble n'est pas du tout favorable à la suppression du Conseil supérieur de la mutualité

Plus précisément, le deuxième alinéa de l'article L. 510-1 du code de la mutualité prévoit qu'il est exercé par le ministre chargé de la mutualité. Il s'avère que ce contrôle n'est pas assuré par le Gouvernement, les mutuelles régies par le livre III étant des organismes de droit privé. Aucun pouvoir de sanction ou d'injonction n'est, à ce titre, conféré à l'État pour rendre cette disposition effective. Le présent amendement reprend donc l'une des recommandations du rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mai 2014, en prévoyant la suppression de l'alinéa précité de l'article

le ministre de la santé n'exerce pas, dans les faits, la compétence de contrôle des mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité. Les activités concernées font l'objet de contrôles par les ARS lorsqu'elles sont réglementées. C'est par exemple le cas pour les établissements sanitaires ou sociaux mutualistes. La commission spéciale a donc souhaité interroger le Gouvernement sur ce sujet, afin de savoir pourquoi le contrôle du ministre de la santé prévu par la loi n'était pas effectif et pour quelles raisons la recommandation formulée en 2013 par l'IGAS n'avait pas été suivie.

une régulation du secteur sans avoir besoin de s'appuyer sur ce conseil. Dans la mesure où l'amendement présenté par Mme Costes vise finalement

15 vise à supprimer le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, le Haut Conseil du dialogue social, la Commission nationale de la négociation

que la volonté du Gouvernement est de favoriser le dialogue social avec les organisations syndicales, quand il ne pense qu'à fusionner

ou évaluation préalable. On ne peut pas nous dire que ces instances ne se réunissent pas. La Comarep, par exemple, se réunit tous les deux mois afin de vérifier notamment la conformité à la loi des accords de branche relatifs à la retraite complémentaire ou à la prévoyance.

qui attendent toujours que l'on prenne en compte leurs demandes et qui se heurtent à un mur. C'est la réalité ! La réforme des

de travail. À défaut d'un réel allégement des procédures administratives de consultation, il permettra une meilleure lisibilité du « paysage » des instances consultatives. Les missions exercées par les diverses instances supprimées continueront d'être assurées. La commission spéciale est favorable au regroupement proposé et s'oppose donc à ces amendements de suppression.

Au-delà du signal négatif ainsi envoyé à toutes les personnes qui s'engagent au quotidien en faveur de l'égalité entre les sexes, cette fusion ne peut qu'entraîner une perte d'expérience et un affaiblissement des outils à disposition des associations féministes.

le Gouvernement va discrètement enterrer l'indépendance d'une organisation qui a démontré toute sa pertinence et son utilité dans les débats publics. Au passage, vous affaiblissez encore davantage les organisations syndicales, qui disposaient grâce à ces instances de moyens pour lutter contre les stéréotypes, la répartition des rôles sociaux et les violences de genre, et pour faire avancer les droits des femmes et la parité en matière politique, administrative et économique, ainsi que dans les domaines de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Telles sont les missions sacrifiées sur l'autel des économies budgétaires, qui seules guident l'action du gouvernement Macron-Philippe. En outre, on demande aux salariés du HCE d'assurer des missions supplémentaires, sans concertation, sans changement de fiches de poste, sans consultation des instances internes, et donc sans avis des organisations syndicales.

la place des femmes dans les conseils d'administration ou encore la négociation collective sur l'égalité, il s'agit de veiller à

La lutte pour l'égalité professionnelle reste une priorité et nécessite l'affirmation d'une ambition politique soutenue et continue, d'autant qu'un effet générationnel semble s'amorcer ; il ne faut pas manquer ce tournant. La disparition d'un organisme paritaire de dialogue social

fusionner le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Quel est l'avis de la commission spéciale ? Aujourd'hui, du fait de lois successives, il existe une instance chargée de contribuer à l'élaboration des politiques publiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de la vie sociale,

Or il ne me semble ni souhaitable ni vraiment possible de traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes en raisonnant en silos, comme si ce que vivent les uns et les autres dans le milieu professionnel était déconnecté de ce qui se passe dans le reste du champ social.

entre les femmes et les hommes dans le recrutement et le déroulement de la carrière des agents publics et privés. Cette préoccupation est prise en compte par les acteurs de la gestion des ressources humaines. Les collectivités territoriales agissent contre les stéréotypes sexistes ou les violences faites aux femmes par la sensibilisation, des actions de communication ou l'organisation d'événements dans les domaines culturel et de l'éducation. Le présent amendement vise à prévoir la représentation de chaque niveau de collectivités territoriales au sein du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'amendement n° 136 rectifié, présenté

ailleurs, s'il fallait définir dans la loi la composition du HCE, il faudrait citer l'ensemble de ses membres. Il serait en effet curieux de ne mentionner que les représentants des collectivités Enfin, je constate que le décret du 3 janvier 2013 fait figurer, parmi les membres du HCE, des représentants des régions, des départements et des communes désignés par les associations d'élus. La commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Or une telle saisine relevait très clairement de l'application du principe de libre administration des collectivités territoriales, et donc du domaine législatif. Par ailleurs, son intérêt résidait notamment dans les échanges entre l'État, les communes et les intercommunalités. La suppression du droit de saisir la commission a privé ces collectivités d'un outil de discussion en amont des projets de documents d'urbanisme. Cet amendement vise à rétablir une version des textes qui ne soit pas en décalage avec la nécessité d'un dialogue entre l'État

par les personnes publiques associées (PPA). Une commune ou un EPCI limitrophe peuvent donc saisir la commission en tant que PPA. Pour ce qui concerne les communes et les EPCI exerçant directement la compétence « urbanisme », leurs rapports sont régis par d'autres règles : l'élaboration des documents d'urbanisme doit intervenir

de l'État, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers et des associations,

permet d'éclairer les élus dans la prise de leurs décisions en matière de documents et d'autorisations d'urbanisme. Elles constituent un outil de lutte contre l'artificialisation des terres agricoles, sachant que la France a perdu un un quart de sa surface agricole ces cinquante dernières années, une situation qui affecte fortement notre résilience alimentaire. Mes chers collègues, ces commissions n'entravent pas les élus dans puisqu'elles émettent essentiellement des avis simples, ce qui est faiblement contraignant. Les avis conformes concernent essentiellement les atteintes substantielles aux productions sous appellation d'origine protégée.

culturel, notamment la protection des salles de spectacle, la labellisation de la création artistique ou encore la reconnaissance des établissements dispensant des enseignements artistiques.

le rôle des collectivités territoriales et la manière d'exercer cette compétence partagée en assurant un égal accès à la culture à tous et sur tout le territoire ? Nous sommes un certain nombre

concerne « la déconcentration des labels artistiques, un mode de régulation financière et de maîtrise budgétaire devra être mis en place, afin d'éviter la constitution d'impasses budgétaires

si les services centraux du ministère de la culture ont vocation à assurer l'équité territoriale, alors ils ont mécaniquement un rôle essentiel à jouer dans la procédure d'attribution et de retrait des labels, et ce rôle va bien au-delà de l'évaluation des diverses structures.

la France porteuse de créations ; la France s'identifiant à un mouvement culturel.

repose sur un socle réglementaire structuré et le périmètre des structures labellisées de la création artistique est largement connu, contrôlé et évalué par les services centraux. L'attribution d'un label à une structure de spectacle vivant ou d'arts plastiques fait l'objet d'un dialogue nourri entre les services centraux et les services déconcentrés, tant pour le respect des critères du cahier des charges et du cahier des missions que du point de vue budgétaire. Le transfert de cette compétence aux préfets de région

Par parallélisme des formes avec les modalités légales d'attribution de ces labels, ce dispositif réglementaire prévoit aujourd'hui que la compétence de retrait revient au ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités et après une période de mise en demeure non respectée. Puisque, nous le savons, le Gouvernement nourrit le projet de donner la compétence d'attribution des labels aux préfets de région, il va de soi que, par cohérence juridique et par parallélisme des formes, il octroiera aussi la compétence de leur suspension ou de leur retrait à ceux-ci. Or, comme c'est Or, comme c'est actuellement ce décret qui règle la question de la suspension du retrait des labels, nous n'aurons pas voix au chapitre- c'est certain -et nous ne pourrons empêcher, comme nous l'avons fait de façon unanime en commission spéciale pour la compétence d'attribution de labels, l'octroi de cette nouvelle compétence de retrait aux préfets. Aussi préférons-nous prévoir, aux termes de la loi et à droit constant, la compétence ministérielle pour mettre en demeure et, éventuellement, pour suspendre ou retirer un label.

est l'avis de la commission spéciale ? Les labels de la création artistique sont au coeur de l'action du ministère de la culture, dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques. Ils constituent des instruments déterminants de sa politique d'irrigation des territoires. Nous pensons qu'il est important que les décisions en matière de label continuent de relever du ministre de la culture ; c'est évidemment un enjeu symbolique pour les structures labellisées,

sans assumer réellement votre politique. C'est d'ailleurs le véritable problème de ce projet de loi. Si vous avez la volonté que, en fin de compte, le ministère de la culture abandonne toutes ses compétences nationales au profit des régions,

aux dépens d'autres régions. Le fait qu'il y ait un ministère de la culture, ayant des compétences nationales, c'est encore la garantie de pouvoir donner à chaque citoyen de notre territoire le même accès à la culture. Un État national, un ministère national cela sert à ça ! Il faut donc que vous nous donniez, aujourd'hui, les garanties que cette mission fondamentale ne sera pas obérée par ce que vous nous proposez. Je n'ai pas entendu, dans votre discours, quelque chose qui nous rassure dans ce domaine. Je

déconcentre les décisions sanitaires du pouvoir politique vers les structures administratives. Pour notre part, nous craignons que, en étendant la compétence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) à un sujet aussi sensible que le contrôle sanitaire des eaux, on ne fasse courir un risque à la santé publique. Si nous avons confiance dans le dévouement et le travail des agents publics, nous connaissons les risques engendrés par les industriels privés,

De la même manière, alors que nous connaissons une pandémie du coronavirus, la gestion des médicaments que les pharmacies internes des hôpitaux peuvent délivrer doit être maintenue aux mains du ministre de la santé. Les transferts de compétences du pouvoir politique aux instances administratives risquent d'entraîner une perte du politique au profit de la technocratie, sur des sujets majeurs. Le transfert du pouvoir politique au profit de la technocratie, qui peut être soumise aux pressions des intérêts privés, nous l'avons malheureusement connue lors de l'affaire du Mediator. toutes ces raisons, nous refusons de reproduire les mêmes erreurs et de déposséder le pouvoir politique des décisions relatives à l'alimentation animale et à la gestion des listes des médicaments des hôpitaux. Quel

du champ « politique » au champ « technocratique ». Le ministre actuellement chargé des agréments visés par l'article 19 exerce précisément ses fonctions comme autorité administrative, ce qui garantit d'ailleurs l'impartialité de ses décisions.

Cette décision sera désormais prise par le directeur général de l'Anses, agence chargée d'instruire les dossiers d'agrément. Or le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève de la compétence de l'État. de l'État. Le droit en vigueur permet de prévenir les situations de conflits d'intérêts. C'est la raison pour laquelle les responsables des laboratoires concernés demandent que la gestion du contrôle sanitaire demeure du ressort de l'État. Tel est l'objet de cet amendement.

en étendant la compétence de l'agence pour agréer des laboratoires, le ministre n'ayant plus qu'un droit d'opposition. Ces dispositions présentent le risque principal de voir agréer un laboratoire en lien direct avec les producteurs et de créer ainsi une situation de conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle les responsables des laboratoires concernés demandent que la gestion du contrôle sanitaire officiel demeure du ressort de l'État. Tel est l'objet de cet amendement. L'amendement n° 197, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi amendement prévoit une exception en maintenant la compétence du ministre chargé de la santé pour la délivrance de l'agrément aux laboratoires réalisant des analyses des paramètres de radioactivité du contrôle sanitaire des eaux. En effet, les missions de l'Anses ne prévoient pas de compétence

Conformément à la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, il faut adapter le niveau de contrainte administrative aux risques que la recherche fait courir aux personnes. personnes. Les recherches non interventionnelles ne font courir, par définition, aucun risque ni aucune contrainte et elles doivent donc faire l'objet de procédures administratives très simples et rapides. grâce à cet amendement, le comité de protection des personnes sera en mesure de délivrer un avis favorable sur l'engagement du promoteur à respecter la réglementation cette évolution permet d'alléger la charge des comités de protection des personnes, ceux-ci pourront dès lors se concentrer sur l'instruction des dossiers les plus à risques et réduire leurs délais de traitement de ces dossiers. Cela permet par ailleurs aux promoteurs de ces recherches de déposer un dossier très simplifié par rapport aux recherches les plus à risques.

Il s'agit de transférer au Comité français d'accréditation les décisions administratives qui relèvent actuellement du groupe interministériel des produits chimiques, en matière de bonnes pratiques de laboratoire.

ont été produits en la matière, le dernier l'ayant été par le Sénat en juin 2019. On consulte partiellement l'ONF. L'étude d'impact est lacunaire sur le contenu de l'ordonnance. L'avis du Conseil d'État ne retient pas la disposition d'habilitation du Gouvernement à modifier le conseil d'administration de l'ONF.

Sur le fond de la réforme, on nous propose une gouvernance centralisée, qui traduit une volonté d'exclusion des corps intermédiaires, notamment les représentants de la filière bois, les associations de protection de l'environnement, mais aussi les collectivités territoriales. Si la commission spéciale a pu apporter une solution sur ce point, ne doit-on pas penser, comme le laissait suggérer le rapport du Comité Action publique 2022, que les forêts communales ne seront plus, à terme, gérées par l'ONF ? On veut également réduire des politiques publiques à des équations comptables. C'est votre spécialité ! On euphémise les difficultés des conditions de travail, qui sont pourtant patentes et qu'accentueront encore la défonctionnarisation et les réductions de personnel. On relègue, bien entendu, les enjeux écologiques et de protection du bien commun. La forêt publique n'est pas un bien économique comme les autres et l'ONF n'est pas une société anonyme qui doit mener une politique commerciale ! Pour 67 % des Français, la forêt est un espace à préserver pour les générations futures. futures. C'est un bien commun. C'est le principal patrimoine public naturel de la France, après le patrimoine maritime, et il est aujourd'hui fragilisé par des menaces climatiques et sanitaires et par la disparition d'espèces. Il faut une structure publique qui dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission d'intérêt général de préservation et de gestion durable de la forêt.

moult services : captage du dioxyde de carbone et, en contrepartie, production du dioxygène nécessaire à notre respiration ; préservation de l'humidité ; protection contre les vagues de chaleur ; régulations de toutes sortes ; espaces-tampons ; protection contre les vents ; lutte contre l'érosion des sols

et mondialisation obligent : insectes ravageurs, plantes invasives, agents pathogènes, incendies ... Nous avons plus que jamais besoin d'un Office national puissant,

la forêt responsable, associant les agents de l'ONF en confiance. Il faut, sans doute, poser le problème sur la table et discuter avec eux. Nous avons besoin d'eux ! Leur expertise nous est précieuse et le sera encore plus dans les années à venir.

bien pensées et, en même temps, un travail intelligent de maintien de la diversité des espèces et de gestion de celles-ci. La filière bois française souffre de fragilités qui sont liées non pas à l'ONF, mais à la structuration des scieries et à d'autres mécanismes. C'est d'ailleurs un point auquel le Gouvernement, au lieu de transformer et de privatiser l'ONF, ferait bien de s'intéresser prioritairement. Nous sommes très hostiles au resserrement du conseil d'administration

n° 34 rectifié . La première disposition de l'article 33 vise à pouvoir faire réaliser par des salariés de droit privé toutes les missions confiées par la loi à l'ONF. Il s'agit de missions de service public administratif, mais aussi de missions de police judiciaire. La réalisation de ces missions essentielles à la protection de la forêt donne lieu à de multiples pressions venant de l'extérieur- acheteurs de bois, usagers, citoyens ... -, mais aussi de l'interne : la situation financière de l'ONF étant chroniquement déficitaire, de nombreuses pressions s'exercent sur les personnels pour augmenter la récolte de bois ou fermer les yeux sur certaines dérives, notamment pour raisons commerciales. Les agents de l'ONF, notamment ceux qui sont chargés de missions de police judiciaire, ont toujours été dotés du statut de fonctionnaire, qu'ils soient en capacité de résister à ces pressions, donc de protéger au mieux forêt et intérêt général, et, d'autre part, pour que la loi soit appliquée en toute impartialité et indépendance. Pour rappel, l'ONF est chargé de protéger et de faire appliquer la loi dans les forêts publiques, qui représentent 10 % du territoire national. Pour remplir ses missions, l'ONF ne dispose plus que de 4 500 fonctionnaires- contre 9 000 en 1985 -, dont environ 3 000 gardes forestiers, répartis sur 10 % de notre pays, de notre pays, outre-mer compris. Ces gardes forestiers travaillent le plus souvent seuls et sont de plus en plus confrontés à la contestation de la puissance publique. Ils représentent, dans de nombreux territoires, une fraction importante, voire majoritaire, des effectifs de police mobilisables en matière de protection de l'environnement et de sécurité publique- d'incendies, de tempêtes, de risques en montagne ... Si les fonctionnaires ne sont pas intrinsèquement plus compétents que des salariés, le statut de fonctionnaire est indispensable pour les agents de l'ONF exerçant ces métiers : pour leur protection d'abord, mais également pour la bonne réalisation de leurs missions, donc pour la protection de la forêt et pour l'intérêt général. Pour ces raisons, le statut de salarié n'est pas adapté à l'exercice de ces missions. Aussi, cet amendement vise à supprimer l'article 33 et, à ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi afin d'élargir les possibilités, pour l'ONF, de recruter des agents contractuels de droit privé.

En deuxième lieu, certaines des évolutions législatives prévues par les habitations sont attendues des acteurs de terrain. S'agissant de l'ONF, tous les travaux conduits ces dernières années, y compris ceux qu'a publiés tout récemment la commission des affaires économiques du Sénat sur la filière bois, convergent sur la nécessité de lui permettre de réformer la gestion de son personnel. Pour ce qui concerne les chambres d'agriculture, le rapprochement des règles applicables aux personnels avec celles que prévoit le code du travail est demandé par Chambres d'agriculture France, auditionnée dans le cadre de nos travaux préparatoires. Enfin, pour répondre aux inquiétudes légitimes soulevées par les auteurs des amendements, la commission spéciale a strictement encadré les habilitations. pour ce qui est de l'ONF, elle a prévu que les missions de police pouvant être confiées à des agents de droit privé soient, d'une part, limitées à la seule constatation des infractions de nature forestière et, d'autre part, exercées par certains d'entre eux, qui sont commissionnés et assermentés à cet effet. Elle a également garanti la présence de l'ensemble des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de l'établissement. S'agissant des chambres d'agriculture, la commission spéciale a prévu le maintien de l'autonomie administrative dont bénéficie le réseau, en prévoyant que le rapprochement des règles puisse être effectué par lui. Elle a aussi veillé à ce que l'évolution statutaire ne se transforme pas en une réforme subreptice du réseau, en indiquant que cette évolution doit intervenir dans le respect de l'organisation et des missions respectives des établissements infranationaux. Enfin, dans les deux cas, la commission spéciale a souhaité que les parties prenantes, organisations syndicales ou collectivités territoriales, soient associées à l'élaboration des ordonnances. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu de supprimer les habilitations à légiférer par ordonnances,

forcément raison à leurs attentes. Je pense en particulier à la représentation des associations de défense de l'environnement, qui peuvent parfois paraître pénibles à certains de nos collègues élus, mais qui sont indispensables à l'équilibre de la gestion de nos forêts. Pour preuve, le Conseil d'État lui-même

il envisage de modifier les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier relatives à la composition du conseil d'administration de l'ONF, lesquelles se bornent à prévoir quatre catégories de membres, le Conseil d'État ne retient pas la disposition l'habilitant à modifier ces dispositions.

M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte (Capam), créée par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance du 20 janvier 2001, par la loi du 21 février 2007 et, enfin, par l'ordonnance du 31 mai 2012. Ce dernier texte, intervenu après la départementalisation de l'île en 2011, prévoyait l'abrogation du régime spécifique de la Capam, au plus tard le 1 janvier 2019, avec pour ambition de replacer Mayotte dans le droit commun. de bricolage en bricolage, de report en report, la Capam, qui avait été imaginée pour s'occuper aussi de la pêche et de l'aquaculture, n'a pu fonctionner que de façon bancale, ces deux secteurs n'ayant, par exemple, jamais bénéficié de dotation.

longtemps. Nous attendons une nouvelle étape, un nouveau souffle, un projet qui ait de la force pour la forêt française. Je suis élu du département qui possède la plus grande forêt domaniale de France.

L'ONF traverse une crise économique et sociale depuis plusieurs années. Le manque d'écoute et de dialogue est au coeur de cette crise. Les syndicats manifestent régulièrement leurs inquiétudes quant à la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Ils rappellent ainsi que l'ONF a perdu 40 % de ses effectifs en trente ans et que cette situation sociale tendue débouche sur une multiplication des suicides. Or le Gouvernement fait ici le choix de réformer par ordonnance, sans permettre au Parlement de s'exprimer sur le fond, ce qui accentuera nécessairement ce sentiment d'opacité. De plus, cette future ordonnance acte le principe de l'élargissement des possibilités de recrutement d'agents contractuels de droit privé à l'ONF. Malgré l'amendement adopté en commission sur l'initiative de Mme la rapporteure, cette mesure inquiète particulièrement les syndicats de l'ONF qui constatent déjà depuis plusieurs années que les instances de l'Office ne recrutent que des agents de droit privé, et non plus des fonctionnaires. Or le statut de fonctionnaire est essentiel pour exercer les missions de police judiciaire, ainsi que l'ensemble des autres missions, de manière impartiale et dans l'intérêt général.

quant à l'élargissement des possibilités de recrutement d'agents contractuels de droit privé au sein de l'ONF. En 2018, le poids des agents recrutés sous statut privé représentait 43 % de la totalité des agents, ce qui est considérable pour un établissement public et interroge sur une atteinte à l'équilibre entre ses missions régaliennes et ses activités concurrentielles. Cette situation interroge également sur l'équilibre entre la préservation des forêts et la gestion productiviste du bois. Le statut de la fonction publique constitue une garantie d'indépendance face aux pressions.

les réalités rencontrées aujourd'hui. Les dispositifs et l'organisation de la filière ne sont pas adaptés aux enjeux et aux impératifs sociétaux qui sont devant nous. La simplification, telle qu'elle est présentée dans cet article 33, aborde le sujet sous un prisme exclusivement administratif et économique, certes important, mais aujourd'hui totalement insuffisant. Pour permettre une réelle efficacité, la gouvernance de l'ONF doit, selon nous, être consolidée dans sa représentativité et donc dans sa légitimité en associant,

en termes de débat et de concertation dans les territoires. Les offices régionaux de la biodiversité constituent des réponses adaptées à la diversité des territoires. Il serait donc également opportun de développer des instances régionales de l'ONF, ouvertes à une gouvernance plus partagée et plus proche des réalités des massifs.

Or la commission spéciale a prévu une solide garantie, en adoptant le principe de la présence de l'ensemble des collectivités territoriales, quel que soit leur échelon, au sein de ce conseil d'administration.

utile. L'amendement n° 30 rectifié est plus problématique. D'une part, son adoption reviendrait à priver le conseil d'administration d'une partie de ses attributions exécutives, alors qu'il est logique qu'un établissement public national tel que l'ONF soit conduit par un organe directorial centralisé. D'autre part, il faut rappeler que l'ONF s'appuie déjà sur des instances en lien avec les territoires : des comités consultatifs, auprès de son conseil d'administration

en rendre compte au Parlement lors du dépôt du projet de loi de ratification. Ces dispositions ayant été introduites par la commission spéciale, en accord avec les acteurs eux-mêmes,

et non dans un comité consultatif annexe, et que cette représentation doit accorder une place aux collectivités propriétaires de forêts relevant du régime forestier. Pour ces raisons, la commission demande le retrait des amendements

il faut réfléchir à une interaction plus forte entre l'ONF et la filière du bois, qui reste profondément défaillante en France. Sur tous ces sujets, monsieur le ministre, il faut une loi d'envergure, une réflexion d'envergure

? Je crains, malheureusement, que les ordonnances et la concertation que vous nous promettez ne règlent que des problèmes techniques, alors que la question fondamentale, elle, sera reportée à un débat ultérieur.

dans le cas de l'ONF, par ordonnances. En commission, notre position n'a pas été majoritaire et les ordonnances ont été maintenues. Toutefois, des aménagements rédactionnels ont été introduits, afin de répondre à certaines inquiétudes.

la durée de l'habilitation, qui est de dix-huit mois, vous envoyez un très mauvais message. S'ils sont satisfaits, maintenez-les ! Cela ne coûte rien et permettrait de rassurer un minimum les organisations syndicales,

Quant à l'amendement visant la décentralisation et les collectivités régionales, là aussi, soyons réalistes ! Nous savons très bien que, demain, pour mieux valoriser nos forêts, nous nous appuierons sur les stratégies locales de développement forestier, qui sont portées par les collectivités territoriales. Si nous voulons être efficaces, nous avons besoin de réactivité et d'une gestion au plus près des massifs.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.